appliquée sur le terrain. L'article 12 du projet de loi prévoit que la rémunération des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par

Si la définition de durées maximales de travail permet de prévenir le risque de surexploitation de la personne détenue et de veiller à sa santé et sa sécurité, celle d'une durée minimale permettrait permettrait d'assurer une garantie de rémunération minimale- même si nous avons bien compris, monsieur le garde des sceaux, que le travail en prison n'était pas très cher payé. Dans le contrat de travail, une règle fondamentale s'impose hors de la prison : celle de la prévisibilité de la durée de travail convenue,

Soilihi, pour présenter l'amendement n° 213 rectifié. L'article 12, nous le savons, s'inscrit dans l'objectif porté par ce projet de loi de redonner du sens à la peine, en favorisant la réinsertion des personnes détenues par la création d'un contrat d'emploi pénitentiaire. L'article renvoie à un décret en Conseil d'État la définition de plusieurs modalités de mise en oeuvre de ce nouveau contrat. Seront notamment définies par ce décret les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif de la personne détenue, ainsi que les conditions dans lesquelles un dispositif d'aménagement du temps de travail, sur une durée supérieure à la semaine, pourrait être mis en place. Lors de l'examen du projet de loi en commission, nos rapporteurs ont apporté une précision pour intégrer le régime des heures complémentaires

aux cotisations retraite. Aujourd'hui, les détenus travaillant en prison sont obligatoirement affiliés à l'assurance vieillesse et peuvent donc acquérir des droits à la retraite.

notamment vis-à-vis des concessionnaires et entreprises extérieures, qui seraient moins enclines à venir offrir du travail aux détenus. Nous attendons de savoir si le Gouvernement prendra des engagements visant

Vivre en milieu carcéral est plus difficile pour les personnes LGBT, en particulier pour les homosexuels et les transsexuels, qui peuvent être victimes de brimades, de harcèlements et de coups. Les femmes transsexuelles incarcérées témoignent être souvent exposées à des propos discriminatoires, de la part tant des autres détenues que du personnel pénitentiaire, peu sensibilisé à la question de la transidentité. Elles sont parfois mises à l'isolement pour leur propre sécurité. Il importe de ne pas nier de telles violences et de faire figurer la lutte contre les discriminations fondées sur l'identité de genre et sur l'orientation sexuelle

à M. Henri Leroy. L'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose que toute personne détenue a droit au respect de sa dignité et de ses droits et que les restrictions liées à la détention tiennent compte de l'âge,

genre ». Ayant, comme d'autres, du mal à comprendre ce drôle de concept, je me suis promené sur la toile. L'identité de genre se définit comme « la conscience que nous avons tous sur le fait d'être homme, femme, ni l'un ni l'autre, ou les deux Il existerait ainsi des agenres, des androgynes, des bispirituels, des cisgenres, des genres fluides, des transgenres, des non-binaires ... J'arrête ici le catalogue. Mes chers collègues, tout cela n'est pas bien sérieux ! Dans notre société, il y a l'homme et il y a la femme. Le rôle du Parlement n'est pas d'importer en France cette novlangue venue tout droit des États-Unis

souhaitait changer la dénomination des avocats généraux à la Cour de cassation, qui n'exercent pas l'action publique et ne sont soumis, selon une coutume séculaire strictement respectée,

de justice par le rapprochement progressif des professions de commissaire-priseur judiciaire et d'huissier de justice. L'ordonnance, dont l'entrée en vigueur est prévue concomitamment à la présente réforme, prévoit néanmoins en son article 25 des mesures transitoires jusqu'au 30 juin 2026.

Nous comprenons le souci de perfection juridique de nos collègues, mais nous pensons que la rédaction adoptée est la plus adaptée au regard de la passion qui a pu exister dans les professions judiciaires sur la question de la composition des juridictions disciplinaires.

préparer les nombreux textes d'application de la réforme de la discipline dans des conditions permettant une réelle concertation des professions. La réforme concerne cinq professions différentes, différentes, qui sont régies par des textes nombreux et épars, comme cela était souligné dans le rapport de l'inspection générale de la justice. Le projet de réforme prévoit des dispositifs nouveaux, qu'il faudra articuler avec les dispositions existantes.

vise à répondre à une inquiétude de la profession d'avocat. En l'état actuel du texte, il y a une forme d'imprescriptibilité des poursuites disciplinaires à l'initiative d'un réclamant tiers à l'encontre des avocats. pourtant un délai de prescription pour les poursuites disciplinaires à l'encontre des officiers ministériels. Nous proposons de limiter dans le temps la possibilité pour un tiers de saisir le bâtonnier. Le délai que nous avons choisi est identique à celui portant sur la responsabilité professionnelle des avocats tel qu'il est défini à l'article 2225 du code civil.

puisse être instruite par le bâtonnier. Lorsqu'à la suite de cette instruction, le bâtonnier décide de n'engager ni poursuite disciplinaire ni procédure de conciliation, deux possibilités s'offrent à l'auteur de la réclamation : saisir soit le procureur général soit directement la juridiction disciplinaire. telle possibilité de saisir directement la juridiction disciplinaire laisse craindre un engorgement de cette juridiction. La question a d'ailleurs été identifiée par le Gouvernement qui indique,

ce filtrage sera assuré par le président de la juridiction disciplinaire. Pourtant, dans sa rédaction actuelle, l'article 28 ne procède à aucun renvoi réglementaire, si bien que l'encadrement de la procédure annoncé par le Gouvernement dans l'étude d'impact ne pourra être suivi d'effet. Faute de garanties apportées par l'exécutif, le présent amendement vise à supprimer la possibilité de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l'auteur de la réclamation, afin de prévenir toute utilisation abusive de la procédure.

conseil de discipline des avocats est une avancée et un progrès pour le droit des clients, et nous ne voyons pas de raison de la supprimer. Contrairement à ce qui a été indiqué, un filtre

28 propose une réforme du régime de discipline des avocats. Il prévoit notamment que toute réclamation déposée à l'encontre d'un avocat puisse être instruite par le bâtonnier. Si celui-ci décide de n'engager ni poursuite disciplinaire ni procédure de conciliation, l'auteur l'auteur de la réclamation peut saisir soit le procureur général soit directement la juridiction disciplinaire. Sans garde-fou, la seconde option laisse craindre un engorgement de la juridiction.

lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l'avocat mis en cause en fait la demande. Cet amendement tend à prévoir que la présidence de ce conseil reste confiée à un avocat, et non à un magistrat, lequel pourra néanmoins, dans l'une des deux situations dérogatoires précitées, participer aux réunions du conseil de discipline en tant que membre. Cela permettrait de continuer à assurer non seulement l'indépendance de la profession d'avocat, mais également l'indépendance entre l'avocature et la magistrature.

parmi lesquels figurent, je le rappelle, les avocats aux conseils, dont la juridiction disciplinaire serait toujours présidée par un magistrat judiciaire, le conseil de discipline des avocats ne serait présidé

le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Par le présent amendement, nous souhaitons

Votre commission a adopté un amendement visant à mieux encadrer la durée de suspension d'un avocat. Il s'agit d'une amélioration des garanties dont bénéficient les avocats. Je ne peux qu'y être favorable sur le principe. Mais, en réalité, cet article est aussi le fondement juridique de la suspension des avocats dans le cadre de la procédure pénale. Compte tenu non seulement de la durée des procédures, mais surtout de l'exercice des voies de recours, il est parfois nécessaire que la suspension puisse se poursuivre au-delà d'un an. C'est d'ailleurs ce qui se passe C'est la raison pour laquelle je vous propose un amendement qui, tout en conservant les avancées de votre commission, tend à permettre la prolongation de la suspension dans le seul cas où une action publique a été engagée contre l'avocat.

J'aurais dû le faire tout à l'heure s'agissant des notaires, mais j'insiste sur celui-ci : l'exemple cité par M. le garde des sceaux n'est pas un cas d'école.

justice d'assister leurs chambres locales respectives dans leur mission de contrôle du respect des obligations prévues en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et, le cas échéant, de sanction.

tel vide juridique a notamment permis le développement de plateformes numériques, souvent scandaleuses, qui jouent sur la frontière très étroite entre l'information et la consultation juridique, afin de réaliser illégalement des prestations juridiques au rabais, et ce au détriment des justiciables et des professionnels du droit. Afin de lutter contre ces braconniers du droit et de protéger l'intérêt du justiciable, nous proposons donc de définir la consultation juridique comme suit une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d'un avis ou d'un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit, en vue, notamment, d'une éventuelle prise de décision. Quel est l'avis de la commission

dans la concurrence entre les avocats et les experts-comptables. C'est pour cette raison que nous aimerions avoir l'avis du Gouvernement. Quel est l'avis du Gouvernement

et de priver les juridictions de leur pouvoir d'appréciation des situations au cas par cas pour s'adapter aux évolutions technologiques. Enfin, je sais bien qu'il s'agit d'une demande récurrente de la profession d'avocat, mais je ne crois pas qu'il soit dans l'intérêt de cette profession d'être enfermée dans une définition

est à Mme le rapporteur. Eu égard aux précisions qui viennent de nous être données par le ministre, je propose à notre collègue de retirer son amendement. Il faut que l'on travaille sur cette définition. Je pense qu'il est intéressant de pouvoir préciser la notion de consultation juridique.

nous nous opposons à ce que certains actes, comme une transaction, un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, contresignés par les avocats des parties et revêtus de la formule exécutoire du greffe, soient reconnus comme des titres exécutoires. L'article s'inscrit dans la continuité des réformes des procédures au civil. Si cette disposition est présentée comme une simplification permettant une accélération des règlements de litiges, il s'agit également d'une déjudiciarisation des procédures. Par ailleurs, la nouvelle procédure prive les parties des garanties inhérentes au contrôle du juge, la vérification n'en étant que formelle. Enfin, cet article ne présente aucun lien avec l'objectif du projet de loi, puisqu'il ne contribue à nos yeux en rien à renforcer la confiance dans l'institution judiciaire. Accélérer les procédures aux dépens de la qualité du contrôle exercé sur celles-ci n'apparaît pas satisfaisant.

serait peut-être inconstitutionnel. En effet, le Conseil constitutionnel permet normalement aux personnes privées d'émettre un titre exécutoire à la seule condition qu'elles soient chargées de l'exécution d'une mission de service public, ce qui n'est pas le cas des avocats.

Nous considérons que c'est une avancée pour les modes alternatifs de règlement des litiges, d'autant que cette préconisation du rapport Perben respecte la jurisprudence du Conseil constitutionnel en conférant aux greffiers

figurait d'ailleurs dans le rapport Perben, permet aux avocats d'explorer un certain nombre de champs nouveaux en matière économique. Ils en ont besoin, parce que c'est une profession durement touchée. Je ne vois pas comment on peut s'y opposer.

L'article 29 du projet de loi ajoute à la liste des titres exécutoires les actes contresignés par avocat dans le cadre des modes amiables de règlement des différends auxquels le greffe a apposé la formule exécutoire. telle disposition a pour objectif de simplifier et de fluidifier les conditions dans lesquelles un accord peut être rendu exécutoire. Toutefois, il ne faut pas que les parties en pâtissent. Or nous avons été sensibles à ce qu'a écrit Mme la Défenseure des droits, Claire Hédon. Dans son avis sur le texte, elle a souligné le risque posé par la rédaction actuelle de l'article au regard de l'information des parties au litige. En effet, l'apposition de la formule exécutoire par le greffe aboutit à éteindre la possibilité de saisir le juge sans pour autant que les signataires de l'accord en soient explicitement avertis. Ainsi, sur la base de ces recommandations de Mme Hédon, le présent amendement vise à sécuriser le dispositif en précisant que la force exécutoire des transactions et des actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative est subordonnée à l'apposition par les parties d'une mention manuscrite prouvant leur connaissance des conditions de la renonciation à l'accès au juge.

pour objet de renforcer l'information des parties en intégrant dans les actes issus des médiations, conciliations et procédures participatives une mention précisant les effets de la renonciation à l'accès à un juge

ou de contestation du fond de l'acte, qui reste de nature contractuelle. Chaque partie sera assistée d'un avocat, à qui il revient de garantir le consentement libre et éclairé des parties aux obligations auxquelles elles

Ce n'est pas parce que la Défenseure des droits écrit un certain nombre de choses que c'est une vérité. C'est sa vérité. D'autres vérités peuvent être différentes.

En pratique, cette extension peut se révéler utile lorsque les parties n'ont pas les moyens de rémunérer un médiateur. Elle est de nature à permettre en toutes circonstances l'effectivité de l'incitation au recours à l'amiable.

à M. Philippe Mouiller. Cet amendement vise, comme en matière familiale, à permettre à tout juge, y compris en référé, de délivrer aux parties une injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur lorsqu'il vide sa saisine, soit pour assurer une bonne exécution de sa décision, soit pour favoriser la recherche d'une voie amiable en mettant à profit le temps qui s'écoulera entre deux instances. C'est le cas par exemple lorsqu'en référé le litige sur le fond n'est pas tranché ou lorsqu'une procédure accélérée au fond ne tranche pas le différend. Il s'agit d'une injonction post-sentencielle ne pouvant qu'avoir des effets bénéfiques pour le traitement de certains contentieux au long cours. ? Madame la rapporteure, Toutefois, ce sont des situations très spécifiques et les généraliser aujourd'hui ne semble pas opportun. L'objet de la médiation est de résoudre un litige. On a l'impression que la mise en place de processus de médiation à l'infini serait quand même contre-productive.

Cet amendement vise à accélérer la mise en oeuvre des mesures de conciliation et de médiation conventionnelle en inscrivant dans la loi que le médiateur ou le conciliateur sont, à l'issue de la séance d'information, en mesure de recueillir l'accord des parties pour entrer en conciliation dès lors que le juge en est informé. Dans la pratique, il est fréquent que les parties souhaitent commencer la médiation aussitôt après avoir reçu l'information sur l'objet et le déroulement de la mesure. l'avis de la commission ? de constater leur conciliation ou leur médiation. Toutefois, seule l'homologation par le juge donne force exécutoire à leur accord. Nous souhaitons en rester là pour le moment.

Il s'agit de donner au juge la possibilité de moduler le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile en fonction du comportement des parties dans la recherche d'une solution amiable, ainsi que des difficultés qu'elles ont rencontrées dans le cadre de ce processus. La rédaction proposée s'inspire de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, qui permet au juge, au stade de la liquidation de l'astreinte, d'apprécier la bonne volonté et les diligences de la personne condamnée à cette astreinte.

Il y a là un déséquilibre, car l'attitude non coopérative peut aussi être imputable à celui qui le perd.

une coordination avec le code civil, afin de permettre aux parties qui ont signé un accord au terme d'une convention de procédure participative, lorsque cet accord est constaté dans un acte contresigné par l'avocat de chacune des parties,

amendement laisse penser qu'il n'y aurait plus le choix pour les parties entre la voie de l'homologation et le règlement amiable. Pour nous, il faut vraiment que les parties puissent continuer à choisir entre la force exécutoire et la voie de l'homologation. C'est pour cette raison que nous sommes défavorables

Maryse Carrère. Cet amendement et les cinq amendements suivants sont issus de la proposition de loi de notre collègue Nathalie Delattre visant à développer le recours à la médiation.

de timides tentatives de développement des procédures de règlement non juridictionnel des différends ont émergé en France, mais aucune politique nationale de l'amiable n'a vu le jour dans notre pays, contrairement à ce qui s'est passé chez nos voisins allemands et italiens notamment. Or la médiation constitue un outil précieux qui permet non seulement de réduire le nombre de jours d'audiencement, mais aussi les besoins matériels et humains nécessaires, le coût des frais de justice supportés par l'État, ainsi que les coûts économiques et sociaux que peut entraîner une rupture brutale des relations entre individus en conflit. En effet, l'intérêt de la médiation est également de permettre aux justiciables de se réapproprier le procès, d'en devenir des acteurs responsables, de porter eux-mêmes leur parole et d'écouter celle de l'autre. Il s'agit de se comprendre mutuellement, d'aborder l'entièreté du conflit, dans ses aspects aussi bien économiques que relationnels, psychologiques ou sociaux. Comment favoriser son développement dans nos procédures judiciaires si la médiation reste un outil flou, mal identifié par nos juges, nos avocats et nos justiciables ? Pour mettre fin à la confusion terminologique autour de ce processus de règlement à l'amiable, l'éclatement des dispositions entre notre code civil et la loi de 1995, notre collègue Nathalie Delattre propose ici un cadre de définition général, en précisant clairement et concrètement le rôle du médiateur.

Carrère. Nous proposons d'introduire le devoir d'impartialité du médiateur et de prémunir celui-ci de tout risque de conflit d'intérêts. Il nous semble primordial que cela puisse être inscrit dans la loi, afin de préserver la sincérité de ce mode de recours à l'amiable.

est à Mme Maryse Carrère. Cet amendement vise à définir les règles de confidentialité dont peuvent bénéficier les parties au cours de la procédure de médiation.

un principe général. Aussi, la confidentialité des échanges apparaît comme un élément nécessaire pour pouvoir poursuivre dans la durée, au-delà du litige, les relations entre les parties. Nous souscrivons tout à fait à cet objectif, mais, là aussi, l'amendement est satisfait, puisque les principes de confidentialité de la médiation sont prévus par l'article 21-3 de la loi

Cet amendement vise à dessiner les contours de la réunion d'information incitant les parties à entrer en médiation conventionnelle ou judiciaire et à prévoir des sanctions pour celles qui ne déféreraient pas à cette injonction du juge.

il convient de garantir la loyauté de chaque démarche de médiation pour l'ensemble des parties. Le médiateur doit en être le garant. Tel est l'objet de cet amendement, qui vise à éviter qu'une partie n'utilise ce recours à l'amiable pour faire traîner un procès en justice.

médiation. Il s'agit d'écarter tout risque pour les parties qui entrent en conciliation ou en médiation conventionnelle avant procès de se voir déclarer irrecevables à agir en justice en raison de l'expiration d'un délai de forclusion que ne suspend pas actuellement la recherche effective d'une solution amiable. cet amendement ne pourra que favoriser le recours à la conciliation ou à la médiation avant saisine du juge, répondant ainsi à l'un des objectifs du projet de loi.

qui est prévu par la loi ou, à défaut, par les jurisprudences. Ces délais ne sont susceptibles ni de suspension ni d'aménagement contractuel. C'est pour cette raison que l'article 2238 du code civil ne suspend que la prescription.

et conseil en propriété industrielle, ou CPI. En effet, si certaines des missions de la profession de conseil sont exercées concurremment ou conjointement avec la profession d'avocat, il apparaît qu'en l'état actuel du droit positif, certaines dispositions législatives fondamentales, notamment sur la garantie de confidentialité, n'offrent pas les mêmes possibilités pour la profession libérale réglementée de CPI que celles dont bénéficient l'avocat, alors même que cette garantie déontologique essentielle pour leurs clients est, dans les faits, la même. Ainsi, il est proposé d'insérer à l'article L. 422-11 la possibilité d'officialiser les correspondances échangées entre un CPI et un confrère ou un CPI et un avocat, sur le même modèle que celui prévu par la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

n'est plus tolérable. Il s'agit, dans la droite ligne de la justice de proximité que je porte, de permettre le développement du réseau d'accès au droit, avec l'appui des juridictions, des professions du droit : provinces, mairies, autorités coutumières et monde associatif.

Avis favorable. Comme l'a indiqué M. le garde des sceaux, cet amendement a fait l'objet d'un travail avec les parlementaires néo-calédoniens, qui y sont très attachés. Je remercie le Gouvernement d'avoir pu permettre l'aboutissement de ces dispositions, levé le gage de l'article 40 et accepté de répondre à cette demande.

Jusqu'à présent, les dispositions relatives à l'aide à l'accès au droit n'avaient toujours pas été étendues à la Nouvelle-Calédonie, ce qui en faisait le seul territoire de la République à ne pas en bénéficier. La création de centres d'accès au droit avait été demandée à l'unanimité du Congrès de Nouvelle-Calédonie dès 2015 et le Conseil d'État avait reconnu la même année la compétence de l'État. Il s'agissait d'une mesure attendue à la fois des institutions calédoniennes et des professionnels de la justice. Le chantier de l'accès aux droits est d'ailleurs un objectif prioritaire dans le plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance 2018-2022, arrêté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Monsieur le garde des sceaux, à l'Assemblée nationale, vous vous étiez engagé devant le député de Nouvelle-Calédonie Philippe Gomès à réparer cette injustice en proposant rapidement une solution. C'est chose faite avec le dépôt de cet amendement, qui est l'aboutissement d'un travail mené de concert, comme vous l'avez rappelé, avec les parlementaires calédoniens Gérard Poadja, Philippe Gomès et Philippe Dunoyer. Nous tenons à vous en remercier. Cette disposition en faveur de l'accès au droit a d'autant plus d'importance dans le contexte référendaire que connaît la Nouvelle-Calédonie.

concernant les signalements adressés par les autorités nationales au procureur européen délégué sur les affaires portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne susceptibles de relever de sa compétence. Cet article 696-11, résultant de la loi du 24 décembre 2020, a en effet prévu des signalements indirects, passant par l'intermédiaire des procureurs de la République spécialisés, sans permettre des signalements directs, notamment par les autorités visées à l'article 40 du code de procédure pénale. Même si ce dispositif est totalement conforme aux exigences du règlement constitutif du Parquet européen, il est cependant souhaitable, dans un souci d'efficacité, comme le demandent le Parquet européen et la Commission européenne, de permettre également des signalements directs, avec simplement une information des procureurs nationaux spécialisés.

eu lieu entre la Commission européenne et d'autres gouvernements quant aux conditions de cette transposition. La proposition qui vous est faite par le Gouvernement vise à permettre la transmission des signalements directement de nos autorités nationales au Parquet européen sans passer par le filtre des parquets. Une telle modification paraît

par l'actuel gouvernement, les ministres s'attribuent des pouvoirs exorbitants sur des sujets qui nécessitent toute l'attention et l'implication des parlementaires. C'est le cas concernant la mise en place de l'interconnexion des casiers judiciaires nationaux par l'article 32 du projet de loi. Cette disposition est loin d'être anodine dont la mise en application est particulièrement délicate et sensible. Nous refusons que les parlementaires soient dessaisis de leurs prérogatives.

M. Henri Leroy. Ce qui est présenté tambour battant comme une révolution est en fait une réforme de coulisses. On attendait que M. Éric Dupond-Moretti garde des sceaux se souvienne des longs réquisitoires que M. Éric Dupond-Moretti avocat dressait contre le système. Le souffle n'est plus le même ! Quelles sont les attentes des Français qui leur permettront de croire de nouveau dans leur justice ? Elles se résument en deux mots

réveillez l'avocat qui sommeille en vous et soutenez cet amendement pour interdire à un magistrat de se syndiquer ! Souvenez-vous de ce terrible épisode du « mur des cons Quel spectacle pitoyable d'un syndicat, le Syndicat de la magistrature, qui se revendique clairement comme organisation de combat ! Hélas ! Ce n'est pas le seul. Il considère la justice et le droit comme des leviers utiles pour obtenir un changement radical de la société. Faute de réaction des autorités politiques de l'époque, cette conception dévoyée du syndicalisme s'est propagée, ce qui a largement participé à saper la confiance des Français dans leur justice. Mes chers collègues, l'incompatibilité avec le statut de magistrat de l'exercice du droit syndical est une nécessité. Elle devrait être aussi naturelle, sinon davantage, que celle des militaires.

un débat a lieu en France pour autoriser les militaires à se syndiquer. Nous sommes favorables à la syndicalisation des militaires qui le souhaitent. Il faut des organisations qui permettent

La crise sanitaire a conduit à mettre en oeuvre de nouvelles modalités de tenue des audiences. Je pense à l'accueil des justiciables, qui étaient parfois empilés dans la même salle. Aujourd'hui, ils sont accueillis séparément, crise sanitaire oblige.

Visioconférence ! Une personne qui sollicite l'ouverture d'une mesure de tutelle au profit d'un parent domicilié dans un autre département est convoquée pour être entendue par le juge des contentieux de la protection ? Visioconférence ! C'est plus fluide, plus proche,

D'abord, la formulation adoptée par la commission présente le risque d'un engorgement que permettrait d'éviter la désignation de plusieurs tribunaux judiciaires, en l'occurrence deux : celui de Paris et celui de Nanterre. Nanterre. Surtout, nous sommes très inquiets des conséquences que pourraient avoir les amendements ayant pour objet la désignation d'un tribunal de commerce dans les affaires relevant du devoir de vigilance. Notre premier point d'inquiétude vient du fait que la définition du devoir de vigilance n'est pas la même selon les juridictions. Les tribunaux de commerce en ont une vision bien plus restrictive. Adopter ces amendements reviendrait à considérer que le devoir de vigilance relève du droit du commerce, donc de litiges relatifs à la gestion interne des entreprises, par exemple sur des enjeux commerciaux entre une entreprise et ses fournisseurs ou, dans ce cas, sur la bonne information par les entreprises de leurs actionnaires sur les risques que présentent leurs activités. Cela reviendrait donc à vider de son sens la loi de 2017 sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre. Puisqu'il semble utile de le rappeler dans cet hémicycle, celle-ci a pour objet d'éviter les violations des droits humains, les préjudices écologiques ou la destruction de l'environnement, la bonne information des actionnaires sur les risques que présentent leurs investissements. Afin de préserver ce mécanisme indispensable qu'est le devoir de vigilance, il est donc inconcevable que les affaires en relevant ne soient pas de la compétence de tribunaux judiciaires. sont les seuls tribunaux à même de juger les entreprises dont la responsabilité pénale est engagée pour de possibles violations de droits fondamentaux. Notre deuxième point d'alerte concerne le fait que l'appel est non suspensif dans les tribunaux de commerce. Si les affaires étaient de la compétence initiale des tribunaux commerciaux, leur renvoi en appel dénué de caractère suspensif ouvrirait donc la voie à la poursuite, pendant des mois, d'activités entraînant des violations graves des droits humains ou des destructions de l'environnement. Dès lors que ces affaires relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, elles entraînent la suspension des activités de l'entreprise, permettant d'éviter des conséquences dramatiques. Ne serait-ce que pour des raisons de cohérence de la loi, nous vous invitons donc à voter cet amendement.

collègue, je souhaite indiquer que réduire le devoir de vigilance à un acte de gestion de l'entreprise à la charge des juges consulaires serait un recul intolérable tant en matière de respect des droits humains que de protection de l'environnement. Les organismes chargés de représenter les intérêts des entreprises, les chambres de commerce et d'industrie par exemple, reconnaissent que les que les tribunaux judiciaires sont mieux équipés pour juger des litiges liés à l'intérêt général. Enfin, nous refusons de nous faire les porte-voix d'entreprises comme Total qui ne respectent pas la loi et tentent de la détricoter en leur faveur. Au contraire, nous proposons de fixer clairement dans la loi le principe selon lequel plusieurs tribunaux judiciaires sont compétents pour juger de ces affaires. Cela constitue un garde-fou indispensable pour assurer l'effectivité du droit de vigilance pour deux raisons : d'une part, cela évite l'engorgement d'une juridiction qui serait unique ; d'autre part, cela met fin aux multiples renvois de compétences entre juges qui allongent les délais de jugement, et ce toujours au détriment des populations gravement touchées par les infractions en cause. L'amendement

compétent pour connaître des actions engagées à l'encontre des entreprises qui méconnaîtraient leurs obligations au titre la loi dite « vigilance », car son expertise et son organisation en font la juridiction la plus compétente pour appréhender une telle mission. La loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre a créé un devoir de vigilance. Il se matérialise notamment par l'obligation pour les sociétés françaises de plus de 5 000 salariés en France ou de 10 000 salariés en France et à l'étranger de réaliser un plan de vigilance. Cette loi dite « vigilance » ne précise cependant pas quel est le tribunal compétent pour connaître des actions engagées à l'encontre des entreprises qui méconnaîtraient leurs obligations. Tel est donc l'objet de l'article 34 du projet de loi, qui vise à attribuer le contentieux du devoir de vigilance à un tribunal judiciaire spécialement désigné. Si la spécialisation des tribunaux s'inscrit dans l'objectif de bonne administration de la justice, il est important de ne pas se tromper de tribunal. Juridiction dotée de compétences en matière économique, mais également de solides connaissances du fonctionnement de l'entreprise, le tribunal de commerce apparaît le mieux placé pour connaître des actions en matière de devoir de vigilance. En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît des contestations relatives à un certain nombre d'engagements. Selon la Cour de cassation, les tribunaux de commerce sont ainsi compétents pour connaître des litiges présentant un « lien direct avec la gestion et connaissent donc déjà des actions en responsabilité civile à l'encontre du dirigeant d'une société. Le plan de vigilance étant inclus dans le rapport de gestion, il est logique que les tribunaux de commerce aient aussi à connaître des actions fondées sur les dispositions des articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce relatives au devoir de vigilance. Confirmant cette analyse, la cour d'appel de Versailles a, dans un arrêt du 10 décembre dernier, reconnu la compétence du tribunal de commerce au motif qu'était « caractérisée l'existence d'un lien direct entre le plan de vigilance, son établissement et sa mise en oeuvre, et la gestion de la société commerciale dans son fonctionnement ». Compte tenu de leur faible nombre et de leur spécificité, il est souhaitable que de tels litiges soient attribués à la compétence du tribunal de commerce de Paris.

une juridiction compétente connaissant le fonctionnement des entreprises- les entreprises mères, les entreprises donneurs d'ordre -et ayant la compétence et la qualification pour apprécier ce contentieux. Nous avions pensé Nous avions pensé au départ que cette spécialisation pouvait relever d'un tribunal judiciaire. Mais, après réflexion et échanges avec nos collègues et de nombreux représentants, nous pensons qu'il est effectivement plus judicieux de conférer cette compétence

pour traiter de ce contentieux du devoir de vigilance, dont les enjeux dépassent parfois largement nos frontières. cohérent pour nous aujourd'hui qu'une telle proposition correspond à la position que défend la commission des lois d'unifier le contentieux économique au sein du tribunal des affaires économiques. Cette position a été défendue

vous avez amorcé un virage très net

mais ce contentieux ne peut pas être celui du tribunal de commerce ! Très bien ! Je sais que le tribunal de commerce a tout fait pour obtenir ce contentieux de façon monopolistique, ce qui me dérange beaucoup.

La compétence du tribunal de commerce doit être écartée dès lors que l'objet des actions engagées sur le fondement des articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce excède largement, largement, voire très largement le seul contentieux du droit des sociétés et de la gestion des entreprises dévolu au tribunal de commerce. Le devoir de vigilance a pour objet de prévenir et de réparer les atteintes graves aux droits humains et aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité des personnes, ainsi qu'à l'environnement.

non le juge du tribunal de commerce. J'ai un respect infini pour les juges consulaires, qui aident notre justice au quotidien, et dans la gratuité et le bénévolat. Mais on ne peut

outre, le dispositif prévu concerne non seulement les plans de vigilance, mais aussi le contentieux de la responsabilité civile, dont le tribunal judiciaire est le juge naturel, rompu à l'exercice juridique consistant à caractériser une faute, un préjudice, un lien de causalité, ainsi qu'à traiter des questions connexes relatives au droit de la preuve ou encore à la prescription. Confier ce contentieux à une juridiction commerciale ne pourrait qu'amener à des distorsions de jurisprudence en matière de droit de la responsabilité civile, génératrices d'une grande insécurité juridique aux dépens des entreprises. Enfin, dans le texte relatif au climat, votre assemblée avait validé la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

présentés. La position du Gouvernement me paraît en cohérence avec les grands principes qui sont les nôtres. Je souhaiterais que le Sénat en revienne

du Rana Plaza au Bangladesh, quand 5 000 personnes sont privées de leurs terres en Ouganda, quand, dans tant de circonstances, des filiales et des filiales de filiales provoquent des dégâts humanitaires

dans des pays souvent très difficiles. Je ne voudrais pas non plus que telle ou telle affaire particulière vînt changer les positions à ce sujet, car c'est toujours le risque.

de parler de « brader » les droits humains aux tribunaux de commerce. Mais je voudrais ajouter des éléments techniques. Si le volume de contentieux venait demain à croître, ce qui n'est pas du tout impossible, la rédaction de la commission se révélerait, on le voit, très contraignante. Elle empêcherait de désigner un deuxième tribunal ou nécessiterait de repasser par la loi pour ce faire.

par une juridiction spécialisée. Nous avons aussi entendu des acteurs du secteur. Si nous soutenons l'amendement de notre collègue Serge Babary, qui est en lien direct avec les entreprises en tant que président de la délégation aux entreprises

de lutter contre les atteintes aux droits garantis par le plan de vigilance, mais en tenant compte de la spécificité du fonctionnement du monde économique et du monde de la concurrence, ainsi que des conséquences pour les entreprises de telles dispositions.

qui a présidé le tribunal de commerce de Marseille, un travail, qu'il a remarquablement accompli, sur les aides aux entrepreneurs qui sont en difficulté ou qui le seront au sortir de la crise. Je n'ai aucune défiance. Mais je trouve franchement qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. D'ailleurs,

beau jeu de nous faire une observation parfaitement exacte. Dans le cadre de l'examen, qui n'est pas très ancien, du projet de loi Climat et résilience, nous avions effectivement donné compétence au tribunal judiciaire ; il ne faut pas le contester.

sujet est, certes, absolument passionnant et a un intérêt juridique, mais il faut en relativiser la portée finale, puisque c'est le même juge qui, dans les deux cas, finira par trancher.

d'avoir accès au fichier des comptes bancaires lorsqu'ils sont porteurs d'un titre exécutoire, alors qu'ils n'ont pas cette faculté dans le cadre d'une ordonnance de saisie conservatoire. Or cela conduit à une distorsion entre notre droit interne et le droit européen dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire, ce dernier étant plus souple en la matière. Nous y trouvons donc une source de discrimination entre les créanciers, selon qu'il s'agisse d'un créancier français ou d'un créancier européen agissant dans le cadre d'une procédure européenne. Aussi, cet amendement tend à modifier la disposition précitée du livre des procédures fiscales, vise à autoriser les huissiers de justice à effectuer une requête Ficoba dans le cadre d'une ordonnance de saisie conservatoire sur comptes bancaires.

à remédier à une rupture d'équilibre injustifiée entre créanciers français et créanciers européens, qui peuvent se prévaloir du règlement sur la saisie conservatoire européenne. Nous souscrivons pleinement à cette démarche et proposons par ce sous-amendement de compléter l'amendement à des fins de coordination avec le code des procédures civiles d'exécution. Nous avions commencé par émettre un avis défavorable sur l'amendement de Mme Carrère lorsqu'est survenu le sous-amendement, pertinent,

Depuis le 1 avril dernier, en vertu de la loi du 23 mars 2019, les huissiers de justice doivent délivrer par voie électronique les saisies attribution et les saisies conservatoires des comptes bancaires. Or les actes adressés par les huissiers de justice font l'objet, dans la plupart des cas, d'un traitement automatique de la part des établissements bancaires. Le taux de rejet est important en raison des difficultés rencontrées par les huissiers au moment de réaliser une saisie, par exemple en cas d'homonymie ou d'erreur dans l'orthographe du nom.

en y ajoutant notamment les dates d'ouverture et de clôture des comptes, ainsi que les numéros des comptes, mais également à leur permettre d'obtenir la date de naissance du débiteur auprès de l'administration fiscale, afin d'améliorer l'efficacité de la procédure.

Historiquement, il s'adressait à l'agence bancaire pour vérifier tel ou tel élément et faire en sorte que la procédure soit techniquement parfaite. Aujourd'hui, il ne peut voir personne, car le processus est informatisé.

qui ont près d'un siècle ont permis de documenter le sujet. Je vous invite à vous référer aux travaux du docteur Magnus Hirschfeld, qui a été l'un des premiers à se pencher sur le sujet.

Je nous y invite d'autant plus que la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, dans un avis tout récent du 25 mai 2021, était très claire sur ce point : « En France, il n'existe [ ...] aucune donnée publique concernant le nombre de personnes transgenres enfermées sur décision administrative ou judiciaire et les études sur les difficultés particulières auxquelles leur transidentité les expose le cas échéant sont embryonnaires. Les pouvoirs publics sont donc dépourvus de données objectives leur permettant d'apprécier efficacement les mesures à mettre en place pour protéger les personnes Dans cette situation, l'élaboration d'un rapport à destination du Parlement paraît indispensable pour que le Gouvernement soit en mesure de protéger, à la fois, ces détenus, mais aussi et surtout la France. Il ne faudrait pas que ces derniers

Si nous demeurons, pour certains d'entre nous, sceptiques quant à la nécessité d'enregistrer et de diffuser les audiences à la télévision, les garanties nouvelles apportées par la commission des lois et nos collègues à l'article 1 nous semblent aussi utiles qu'importantes. Par ailleurs, nous souscrivons pleinement à l'encadrement dans le temps de la durée de l'enquête préliminaire, tout comme au renforcement des garanties qui protègent le secret professionnel des avocats. Nous saluons la suppression de l'article 5, qui tendait à limiter le placement en détention provisoire, la prolongation de l'expérimentation des cours criminelles départementales jusqu'en 2023, ainsi que le remplacement du rappel à la loi par le nouvel avertissement pénal probatoire tel qu'amendé par le Sénat. groupe se félicite également de l'inscription dans le texte du Sénat de l'amendement, adopté ici avec une réelle émotion sur l'ensemble des travées, autorisant la révision des condamnations pénales prononcées sous l'empire du code d'instruction criminelle après usage de la torture, en écho à l'affaire Mis et Thiennot, dans le département de l'Indre. Nous regrettons évidemment que plusieurs amendements de nos collègues Les Républicains n'aient pas pu être adoptés. Néanmoins, il nous semble malgré tout que le texte voté ce soir par le Sénat apporte un certain nombre de garanties supplémentaires au projet de loi de M. le garde des sceaux et traduit la force des convictions de notre assemblée. Nous espérons que le dialogue constructif du Sénat avec les acteurs du monde judiciaire, à l'image de celui conduit avant-hier lors de l'Agora de la justice animée par le président Gérard Larcher, ainsi que la richesse des travaux de fond menés par la commission des lois, en plus de l'adoption de ce projet de loi, permettront de renforcer un peu plus la confiance dans la justice de nos concitoyens. nos concitoyens. Je voudrais remercier très chaleureusement les rapporteurs Agnès Canayer et Philippe Bonnecarrère de la qualité de leur travail, sous la présidence attentive et expérimentée du président de la commission des lois, François-Noël Buffet.

des cours criminelles départementales, Thani Mohamed Soilihi. Notre amendement vise, dans un souci de cohérence, à ajouter aux compétences des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles l'ensemble des compétences de magistrats exerçant à titre temporaire. Les magistrats honoraires sont d'anciens magistrats de carrière, déjà essentiel pour les juridictions. L'extension de leurs compétences se justifie donc pleinement, d'autant qu'elle permettra de dynamiser et de diversifier les candidatures à ces fonctions, ainsi que d'offrir une plus grande souplesse aux juridictions.

puisque nous souhaitons l'élargissement des compétences des magistrats honoraires et leur alignement sur celles des magistrats à titre temporaire.

exerçant à titre temporaire dont l'expérience professionnelle antérieure garantit une excellente connaissance des fonctions judiciaires. Cette dispense s'appliquera évidemment aux avocats honoraires.

Et la Convention européenne prévoit que des restrictions légitimes puissent être opposées à l'exercice du droit de se syndiquer pour certaines catégories de fonctionnaires. Le code de la défense a été réformé en conséquence pour maintenir cette interdiction tout en la tempérant.

de la commission, modifié, l'ensemble du projet de loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire